La séance est reprise. M. le président du Sénat a été informé par M. le Premier ministre, par lettre en date de ce jour, en application de l'article 35, deuxième alinéa, de la Constitution, que le Gouvernement a décidé de faire intervenir nos forces armées au Tchad contre des groupes armés venus de Libye, en réponse à la demande d'assistance des autorités tchadiennes formulée par le Président de la République du Tchad, M. ldriss Déby Itno. Itno. M. le Premier ministre a demandé à Mme la ministre des armées de tenir le Parlement informé de l'évolution de la situation. Acte est donné de cette communication. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises. Nous poursuivons la discussion de l'article

Imposer un mécanisme de lien obligatoire entre intéressement et plan d'épargne d'entreprise rend complexe une mesure simple. Laissons l'employeur libre, en cas d'accord d'intéressement, d'ouvrir ou non un PEE pour ses salariés ! Tel est le sens de cet amendement de rétablissement. L'amendement

: je pense au contraire qu'il faut donner au salarié le choix de l'orientation de son épargne. Cela me semble extrêmement important. Pourquoi obliger le salarié à percevoir tout de suite son épargne s'il souhaite la placer sur le moyen terme ?

amendement vise à sécuriser les exonérations offertes pour les accords d'intéressement tout en laissant à l'administration le temps nécessaire pour analyser ces accords. Nous partageons l'objectif de M. le rapporteur : apporter une plus grande sécurité juridique aux accords d'intéressement une fois ceux-ci signés et déposés à la DIRECCTE. Le droit actuel prévoit d'ores et déjà une sécurisation des sommes versées vis-à-vis des URSSAF, pour l'année en cours et, le cas échéant, Le texte de la commission va plus loin en permettant une sécurisation du traitement social pour la durée restante de l'accord. Toutefois, le contrôle de légalité des accords d'intéressement doit pouvoir s'opérer dans un délai suffisamment raisonnable pour garantir la conformité de l'accord à la loi.

les résultats comptables de l'année pour pouvoir déterminer si l'accord d'intéressement a été atteint. En réalité, un délai de huit mois laisse largement le temps à l'exercice de se faire. C'est l'expérience que j'en ai en tant que chef d'entreprise.

: La parole est à M. Martin Lévrier. Cet amendement de rétablissement vise à ne pas autoriser les entreprises, lors de la conclusion d'un premier accord d'intéressement, à conclure cet accord à tout moment de l'année en contrepartie d'une extension à quatre ans de la durée de l'accord. En effet, afin de respecter le caractère aléatoire de l'intéressement, l'accord doit actuellement être conclu au cours du premier semestre de l'exercice. Une conclusion trop tardive de l'accord pourrait remettre en cause le caractère aléatoire de la formule d'intéressement et fragiliser juridiquement l'accord dans les faits. Si l'entreprise souhaite conclure un accord et verser de l'intéressement au cours du même exercice, elle peut opter pour une période de calcul infra-annuelle, ou verser des acomptes, à condition que l'accord le prévoie.

les entreprises puissent éventuellement souscrire un accord d'intéressement au-delà du 30 juin, qui est aujourd'hui la date limite, tout simplement parce que les discussions se prolongent parfois un petit peu.

Il nous paraît dommage d'exclure de ce système toutes les entreprises comptant moins de 50 salariés. Nous proposons donc de ramener le seuil à 10 salariés. D'autres amendements tendent à proposer un seuil de 20 salariés, mais ce choix ne nous paraît pas cohérent. Le seuil de 20 salariés a été conservé exclusivement dans la loi pour les travailleurs en situation de handicap. Dans un souci de simplification, il nous paraît plus intelligent d'utiliser les seuils essentiels et pas le seuil exceptionnel de 20, d'où notre proposition de ramener ce seuil à 10 salariés Quel

n° 167 rectifié. L'article 57 supprime la possibilité d'affecter les sommes constituant la réserve spéciale de participation à un compte courant bloqué géré par l'entreprise. Cette disposition, introduite en commission spéciale, vise à protéger les salariés contre un investissement risqué par rapport aux autres méthodes d'affectation de la participation. S'il est vrai que, dans les entreprises dites classiques, ce dispositif est peu utilisé et peut paraître asymétrique dans son rapport de force, il en est autrement dans les SCOP, où, par définition, les salariés sont les associés de l'entreprise. Dans les SCOP, le recours au compte courant bloqué n'est pas un risque pris par les salariés pour leur épargne, c'est un investissement volontaire de leur part dans la trésorerie de l'entreprise qu'ils gèrent et contrôlent. C'est pourquoi le présent amendement vise à conserver la possibilité d'affectation à un compte courant bloqué uniquement pour ces dernières. Si les SCOP ont prouvé leur durabilité, avec un taux de pérennité à cinq de 67 %, c'est notamment parce qu'elles peuvent compter sur l'investissement de leurs salariés, associés de l'entreprise. Pour assurer leurs besoins en trésorerie, certains salariés des coopératives préfèrent en effet verser leur part de la réserve spéciale de participation sur des comptes courants bloqués plutôt que de la récupérer par versement direct ou de l'épargner dans un dispositif financier qui ne bénéficiera pas à l'entreprise. Aussi, supprimer le versement de la réserve spéciale de participation sur un compte courant bloqué priverait les SCOP d'un des outils qui assure aujourd'hui leur succès,

puisque les salariés sont partie prenante des décisions prises. Les comptes courants ne peuvent être affectés qu'à l'activité de l'entreprise. Les priver de cette opportunité,

à adapter les mécanismes proposés aux spécificités de l'économie sociale et solidaire ? Monsieur le rapporteur, je comprends votre souci de simplification, mais, simplifier, ce n'est pas uniformiser ! Simplifier pour les acteurs concernés, c'est moins de bureaucratie, moins de complexité, moins d'incompréhension par rapport au dispositif. Ce dispositif n'a jamais été contesté par quiconque dans le monde coopératif.

Or la formulation retenue « sans qu'ils puissent excéder le produit financier du placement » peut poser problème. Si les produits financiers sont négatifs, on pourrait imaginer des frais financiers négatifs. Afin d'éviter ce genre d'incompréhension, nous proposons que le niveau des plafonds pour les frais de tenue de compte reste simplement fixé par décret.

l'amendement n° 993. Tel que rédigé, l'encadrement des frais de gestion du PERCO prévu par le texte issu de la commission spéciale peut sembler dysfonctionnel. Il pourrait conduire à des frais de gestion négatifs dans l'hypothèse où les produits financiers auraient un rendement négatif. La rédaction de l'amendement n°

ambiguë. En effet, elle donne un caractère obligatoire à la négociation dans les branches professionnelles d'un accord sur « un régime d'intéressement, de participation ou d'épargne salariale » en précisant qu'il « est adapté aux entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche et que « les entreprises de la branche peuvent opter pour l'application de l'accord ainsi négocié ». On pourrait donc penser, par ricochet, que les dispositifs relatifs à l'intéressement et à l'épargne salariale deviennent obligatoires, notamment pour les entreprises de moins de 50 salariés- l'entreprise ayant le choix entre les dispositions résultant d'un accord conclu son sein et les dispositions prévues dans l'accord de branche -, alors que ces dispositifs, en particulier l'intéressement, sont créés sur la stricte base du volontariat. La rédaction proposée dans le présent amendement vise à éviter toute ambiguïté. Elle rappelle à la fois le caractère facultatif de la mise en place de dispositifs d'intéressement et d'épargne salariale et précise le caractère purement volontaire

à M. Jean-Marc Gabouty. L'équité fiscale, le partage des richesses, le pouvoir d'achat sont des enjeux majeurs pour notre cohésion sociale. Ces attentes ressortent très largement en tête des réunions organisées dans le cadre du grand débat national. L'élargissement du champ d'application de l'intéressement peut contribuer à répondre à ces attentes. Cet amendement vise à rendre obligatoire l'intéressement dans toutes les entreprises de plus de 10 salariés qui n'ont pas mis en place un accord de participation. L'intéressement est peu utilisé dans les PME sur la base du volontariat. C'est pourtant un dispositif simple, concret et facile à mettre en oeuvre, y compris dans les petites entreprises : cela fait trente ans que je le pratique. Les modalités de calcul du plancher, du plafond ou de la base peuvent être fixées ou améliorées par décret, ce qui laisse au Gouvernement la faculté d'adapter au mieux ce dispositif. Cette application obligatoire de l'intéressement aux PME est à la fois dans l'intérêt des salariés et dans celui des entreprises. Il génère plus de justice, il améliore la rémunération, il favorise des négociations salariales plus apaisées et il augmente la motivation des salariés dans la recherche de performances et de résultats. Le gage vise à compenser la perte de recettes au titre de l'impôt sur les sociétés, qui doit être en contrepartie équilibré par une hausse des recettes au titre de l'impôt sur le revenu et de la TVA par un surplus de consommation.

relevant le seuil de 50 à 100 salariés vous privez les salariés des entreprises de cette tranche de la garantie de bénéficier de la participation, qui passe ainsi sous régime optionnel. Cela ne me paraît pas vraiment être un progrès. Cet amendement tend à compenser les effets pervers de ce relèvement de seuil. vaut aussi pour le Gouvernement si les propos de M. le ministre sur un éventuel relèvement à 70 du seuil de 50 venaient à être mis en oeuvre ... La position que j'exprime est éminemment politique. Je la soumets à votre approbation dans un contexte social qui demande un peu de courage, sinon de l'audace

nos yeux, l'intéressement est par nature un dispositif collectif négocié avec les salariés et facultatif. Cet amendement rendrait obligatoire l'intéressement dans les entreprises de plus de 10 salariés et de moins de 50. Cette mesure risque d'introduire une confusion entre deux dispositifs- l'intéressement et la participation -et d'alimenter l'idée qu'il conviendrait de les fusionner. Il nous apparaît essentiel de conserver les deux instruments, qui visent des objectifs distincts. L'intéressement permet notamment d'avoir une certaine liberté quant à la fixation

creusés éventuellement par l'exercice précédent. Je souhaite donc donner la possibilité de reporter dans la base de calcul, lorsqu'elle a un caractère financier, le résultat de l'année précédente. Je précise que le résultat doit être le même résultat de référence- le bénéfice net comptable, par exemple, ou le bénéfice d'exploitation -de manière à lisser

Quel est l'avis du Gouvernement ? L'employeur et les représentants du personnel disposent d'ores et déjà d'une certaine marge de manoeuvre afin de déterminer la formule d'intéressement la plus adaptée pour encourager la participation des salariés. L'ajout explicite dans le code du travail de la prise en compte du résultat comptable de l'exercice précédent, si celui-ci est négatif, nous paraît quelque peu surcontraindre le dispositif, ce qui n'empêche pas de tenir compte du cycle dans lequel se trouve l'entreprise et d'avoir une approche pluriannuelle. L'avis est donc défavorable.

M. Jean-Louis Tourenne. Cet amendement vise à mettre en place une procédure de déclaration dématérialisée et pré-remplie pour les entreprises de moins de 50 salariés, afin d'y faciliter la diffusion des dispositifs d'épargne salariale. Cette déclaration comporterait l'ensemble des mentions obligatoires prévues à l'article L. 3313-2 du code du travail, simplifiant ainsi le contrôle par l'administration. Elle allégera et simplifiera également les démarches des PME pour offrir une épargne salariale à leurs employés.

Tourenne. La réserve spéciale de participation est calculée selon une formule tout à fait particulière et compliquée : il faut multiplier un coefficient d'un demi par le résultat fiscal, duquel on retire 5 % des capitaux propres pour assurer la rémunération des capitaux. On multiplie enfin ce résultat par le montant des salaires sur la valeur ajoutée.

et de lisibilité des dispositifs d'intéressement et de participation, parce que je considère que c'est la clé de leur réussite. Si les interlocuteurs concernés, qu'ils soient chefs d'entreprise ou salariés, ne comprennent pas

C'est une participation aux résultats de l'entreprise, ce n'est pas une charge ! Il s'agit d'une juste répartition entre ceux qui font la richesse de l'entreprise et ceux qui en sont,

Le plafond annuel de la sécurité sociale, le PASS, a été fixé à 40 524 euros par an. Cette valeur a une incidence fiscale : elle sert à calculer le plafond de déduction du revenu applicable aux dispositifs d'épargne salariale et d'épargne retraite. Le présent amendement vise à abaisser le plafond du salaire pris en compte dans le calcul de la redistribution proportionnelle de la participation à deux PASS, contre trois actuellement. L'effet sera mécanique : ceux qui perçoivent plus de deux PASS percevront un peu moins d'intéressement, au bénéfice de ceux qui sont en deçà de ce nouveau plafond et qui pourront percevoir jusqu'à 80 euros de plus par an. Au sein d'une même entreprise, demander cet acte d'entraide aux employés dont le salaire est supérieur à 6 750 euros par mois me semble être un geste d'équité. La parole

à récompenser la performance des salariés, mais à leur faire bénéficier des résultats de l'activité à laquelle ils contribuent. Dans le contexte social tendu que nous connaissons depuis plusieurs mois, cette mesure de justice salariale peut apparaître comme une réponse, parmi d'autres,

Je tiens à rappeler que l'employeur doit demander l'adresse du salarié quittant son entreprise avant le versement des primes de participation ; en contrepartie, le salarié doit l'aviser de tous ses changements d'adresse. S'il ne peut S'il ne peut être contacté à l'adresse connue, les avoirs doivent être tenus à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite du versement. Passé ces délais, ces avoirs doivent être versés à la Caisse des dépôts et consignations. Le premier point de l'amendement viendrait modifier ce processus, mettant ainsi en péril la possibilité pour les salariés de récupérer leur avoir. Il instaurerait, en second lieu, une rupture d'égalité entre les salariés, puisque seuls ceux des entreprises de travail temporaire pourraient se voir opposer une condition d'ancienneté de six mois.

est l'avis du Gouvernement ? Cet amendement vise à supprimer un article qui permet aux salariés d'entreprises non cotées de débloquer leur plan d'épargne de manière anticipée pour investir dans l'acquisition de parts sociales de leur entreprise. La suppression proposée ne paraît pas souhaitable : l'article 57 permet en effet de développer l'actionnariat salarié, ce qui est l'objectif du projet de loi PACTE, et aux salariés des entreprises non cotées d'avoir accès à l'actionnariat dans les mêmes conditions que les salariés appartenant à des sociétés en actions. donc de rétablir un équilibre. Par ailleurs, les réserves exprimées, notamment du point de vue de la stabilité juridique des SARL, doivent être relativisées, car l'article 57 n'introduit pas de droits nouveaux à l'actionnariat et ne contredit en rien le statut des SARL.

Pour ce faire, l'amendement vise à préciser les mentions que devra contenir le décret auquel les teneurs de comptes feront référence pour éditer le relevé d'informations relatif au plan d'épargne des salariés. salariés. L'article ainsi amendé disposera que le décret applicable au relevé contient, en plus de la date d'édition du relevé, les versements et retraits effectués l'année précédente sur le plan d'épargne.

actions gratuites ! C'est ce qu'ont reçu, fin septembre, 25 000 employés de chez Alstom dans le cadre de son plan d'actionnariat salarié mis en place en 2016, soit un gain de 1 200 euros brut par tête. La France est championne européenne en matière d'actionnariat salarié : la part du capital des sociétés cotées détenue par les « collaborateurs » y est de 4 %, contre 1,6 % pour la moyenne européenne. Au total, ils seraient 3,5 millions à avoir franchi le pas dans Pour notre part, si nous n'avons pas d'allergie idéologique, nous ne défendons pas l'actionnariat salarié : lorsque l'on place son argent, il ne faut pas mettre ses oeufs dans le même panier. Or, en choisissant un tel placement non diversifié, le salarié expose son épargne et son travail au même risque. Chez Areva, le dispositif n'a pas fait que des heureux. En 2015, deux ans après avoir acheté des actions, les salariés ont vu la valeur de celles-ci fondre de près de la moitié. Plusieurs d'entre eux ont déposé plainte pour « délit de fausse information », estimant que leur direction leur avait caché les mauvais résultats de l'entreprise pour les inciter à acheter des actions. Au sein du groupe Orange, qui a mis en place un dispositif d'actionnariat salarié dès 1997, lors de la privatisation de l'entreprise, l'aventure n'a guère été plus reluisante. Le cours d'introduction à l'époque était de 28 euros ; aujourd'hui, il tourne autour de 14 ou 15 euros. L'actionnariat salarié n'améliore en rien les rémunérations. Pis, il s'accompagne toujours d'une modération salariale. C'est un dispositif en réalité tourné vers des objectifs financiers, avec une logique managériale incitant les salariés à être toujours plus productifs. Pour les employeurs, cela permet surtout de transformer une charge d'entreprise en fonds propres, au lieu de mettre en place d'autres dispositifs sur la rémunération qui ont coût immédiat. C'est une politique sociale à moindres frais. La représentation syndicale dans les conseils d'administration est un bien maigre avantage face à l'ensemble de ces régressions. Nous demandons la suppression de cet article, car, si les rémunérations des travailleurs sont trop basses, il est nécessaire de revaloriser les salaires plutôt que de passer par des systèmes de rémunération de substitution. Quel est l'avis de la commission spéciale ?

il s'agit de permettre aux salariés de devenir actionnaires. On ne peut pas être contre ce principe ! Si ! Les salariés sont forcément intéressés à la bonne marche de leur entreprise.

est un attachement à l'entreprise s'exerçant par le biais de l'actionnariat d'entreprise. On ne répartit pas autre chose que des parts de l'entreprise en faisant cela, alors pourquoi l'empêcher ? Je ne comprends pas ! Certes, c'est

faisons en sorte que les salariés aient un bon pouvoir d'achat

Bah alors ? Ma chère collègue, un peu de patience, j'en arrive à ma démonstration. Pour les patrons, l'épargne salariale, par le jeu des exonérations de cotisations sociales, 40 % moins cher qu'une augmentation de salaire. Cela devrait nous faire réfléchir, nous qui sommes toutes et tous d'accord pour l'augmentation des salaires, lesquels nous semblent insuffisants. L'épargne salariale fait dépendre la rémunération des salariés des profits de l'entreprise ou de l'évolution du cours des actions en bourse. C'est cette logique

Ceux qui siègent dans les différents comités, directoires et comités de direction peuvent représenter une partie importante des salariés. Ils ont donc un poids certain dans la prise de décision. C'est ainsi que je vois

et reconnaître ainsi que la plus-value produite tient largement à la contribution de ces salariés. Cet amendement prévoit ainsi la formalisation sur une base volontaire d'un accord entre l'investisseur et l'entreprise dans laquelle il investit, par lequel celui-ci s'engagerait à reverser une fraction de la plus-value au terme de la période d'investissement. L'entreprise serait chargée de redistribuer ces sommes aux salariés ou anciens salariés au prorata de leur durée de présence dans l'entreprise. D'un point de vue fiscalo-social, les sommes versées s'apparenteraient à un abondement unilatéral de l'employeur sur le plan d'épargne d'entreprise, qui jouit du même traitement fiscalo-social que l'intéressement forfait social pour l'employeur, défiscalisation pour le salarié dans la limite du plafond de droit commun. Les sommes seraient également soumises au forfait social, qui serait directement déduit par l'entreprise des sommes versées pour le compte de l'investisseur, de sorte qu'aucune charge nouvelle ne pèserait sur elle. Des mesures de coordination fiscale sont également prévues pour éviter toute double imposition des sommes ainsi versées. Ce dispositif permettra de développer le partage de la valeur au profit des salariés dans l'industrie de la gestion d'actifs, en particulier dans des opérations où, comme vous le savez,

parole est à Mme la secrétaire d'État. On parle de l'OCDE, mais, comme nous sommes au sein d'une chambre du Parlement français, je citerai une note du Trésor qui reprend le rapport de l'OCDE : « La part du travail dans la valeur ajoutée a reculé depuis les années 1990 dans la plupart des grands pays de l'OCDE au profit généralement d'une amélioration du taux de marge, sauf en France.

des dépenses sociales mondiales. Ce n'est pas vraiment un modèle apparemment ... Dans d'autres pays, c'est l'accumulation de capital, autrement dit l'épargne, qui permet l'investissement et donc le travail. Voilà une piste pour faire baisser le chômage

Cet amendement a pour objet de permettre aux fonds communs de placement d'entreprise de détenir des parts d'une société coopérative. Aujourd'hui, les parts sociales des banques coopératives et des coopératives dans leur ensemble sont des actifs spécifiques qui ne sont pas éligibles à un FCPE. Par conséquent, alors que les salariés d'entreprises de droit privé peuvent détenir des actions de leur entreprise en épargne salariale, les salariés des entreprises coopératives sont privés de cette faculté. À cette observation, la commission spéciale m'a répondu que cet amendement était satisfait par le droit existant.

du Gouvernement ? J'ai la même analyse technique sur les articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier. Si je comprends bien, les schémas existants de FCPE confirment la faisabilité actuelle de ce dispositif.

Le dispositif d'actions gratuites avait été inscrit dans la loi Macron de 2015. Il avait pour objectif de permettre à un créateur d'entreprise n'ayant pas les moyens de recruter un ingénieur, par exemple, de lui attribuer des actions gratuites afin de l'intéresser au développement de la société. Initialement, l'esprit qui a présidé à la création de ce dispositif était de permettre aux petites entreprises d'être plus attractives pour leurs salariés. Cet esprit a été dévoyé, puisque le dispositif a été étendu à toutes les entreprises du CAC 40, pour lesquelles la logique, vous en conviendrez, est bien différente. En effet, ces entreprises disposent de moyens suffisants, qu'elles peuvent parfaitement mettre en oeuvre afin d'attirer les salariés. Elles n'ont pas besoin de bénéficier d'un allégement de la contribution, contrairement aux petites et moyennes entreprises. Dans le cadre de la loi de finances rectificative de 2016, un taux de 30 % avait été fixé pour les grandes entreprises,

je suis déjà intervenue sur la question. Nous nous opposons à ces décisions successives qui vident progressivement les caisses de la sécurité sociale, comme en attestent les chiffres que nous vous avons fournis, quoi que vous en disiez, madame la secrétaire Puisque cette section du projet de loi a pour objet de rendre les entreprises plus justes et d'assurer un meilleur partage de la valeur, il ne nous paraît que justice que les entreprises continuent de participer à notre système de solidarité nationale à hauteur de leurs moyens. C'est pourquoi nous vous proposons de rétablir le taux de 30 % de la contribution applicable

le conseil débat des performances des dirigeants mandataires sociaux exécutifs, hors la présence des intéressés. « La détermination de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux exécutifs relève de la responsabilité du conseil d'administration qui les nomme et se fonde sur les propositions du comité des rémunérations. Le conseil motive ses décisions prises en la matière. « La rémunération de ces dirigeants doit être compétitive, adaptée à la stratégie et au contexte de l'entreprise et doit notamment avoir pour objectif de promouvoir sa performance et sa compétitivité sur le moyen et long terme en intégrant un ou plusieurs critères liés à la responsabilité sociale et environnementale. « La rémunération doit permettre d'attirer, de retenir et de motiver des dirigeants performants. « Le conseil peut décider d'attribuer une rémunération variable annuelle dont le paiement peut, le cas échéant, être différé. « Les règles de fixation de cette rémunération doivent être cohérentes avec l'évaluation faite annuellement des performances des dirigeants mandataires sociaux exécutifs et avec la stratégie de l'entreprise. Elles dépendent de la performance du dirigeant et du progrès réalisé par l'entreprise. Les modalités de la rémunération variable annuelle doivent être intelligibles pour l'actionnaire et donner lieu chaque année à une information claire et exhaustive dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise. Le conseil définit les critères permettant de déterminer la rémunération variable annuelle ainsi que les objectifs à atteindre. Ceux-ci doivent être précis et bien entendu préétablis. Il doit être procédé à un réexamen régulier de ces critères dont il faut éviter les révisions trop fréquentes. » À la vérité, ce code se substitue, dans les faits, à la moindre disposition tendant à réduire ou encadrer la rémunération des dirigeants d'entreprise. Tout, dans ce code de gouvernance, fait de chaque situation un cas d'espèce, uniquement résolu par les décisions du conseil d'administration de l'entreprise, où, de manière générale, on peut coopter ceux qui sont, ailleurs, en situation de dirigeant salarié. Sans autre règle que celle de la décision interne de l'aréopage des dirigeants de l'entreprise, nous aboutissons aux situations excessives maintes fois dénoncées et dont l'affaire Ghosn est une sorte de point d'orgue. C'est donc pour poser des règles claires de salubrité publique et sociale que nous vous invitons à adopter cet amendement. Quel

Je ne comprends pas du tout cet amendement, qui vise la rémunération des administrateurs et des membres du conseil de surveillance.

puisque les actions remises aux bénéficiaires sont des actions existantes rachetées par la société. De telles attributions n'étant pas dilutives, une autorisation par une assemblée générale extraordinaire ne se justifie pas. Il est rappelé que, par l'ordonnance du 31 juillet 2014, la compétence pour décider de l'émission de valeurs mobilières non dilutives, comme les obligations convertibles en actions existantes, a été transférée de l'assemblée générale extraordinaire vers le conseil d'administration de la société émettrice. De la même manière, les conditions d'autorisation des attributions d'options d'achat d'actions existantes pourraient être allégées, favorisant ainsi le développement de l'actionnariat salarié. Quel est l'avis de la

du Gouvernement ? La compétence de l'assemblée générale extraordinaire est justifiée dans toutes les opérations d'accès au capital. Vous avez raison de distinguer les attributions

au sein de la même société, notamment les agréments en cas de regroupement des actions de plusieurs actionnaires dans une société civile en participation, relève non pas de l'assemblée générale extraordinaire, mais de l'assemblée générale ordinaire.

de vous vous faire part d'une curiosité concernant les conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise, les FCPE,

comprennent deux tiers de salariés : « En 2017, plus de 2 millions de salariés sur les 4,2 millions ayant versé dans un fonds d'épargne salariale l'ont fait dans un fonds disposant d'une gouvernance, avec au moins deux tiers de salariés parmi les administrateurs.

en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité, ainsi que la définition de leur raison d'être. En complétant deux articles du code civil, cet article fait peser un risque juridique et contentieux important sur les sociétés de toute taille. En effet, ce texte est de nature à favoriser des actions en responsabilité liées à la prise en considération, que certains acteurs pourraient estimer insuffisante, des enjeux sociaux et environnementaux. Comment le juge interprétera-t-il la notion imprécise de prise en considération de ces enjeux ? Aussi, dans le but de ne pas fragiliser les entreprises, notamment les moins grandes,

dans les entreprises ou les organisations représentatives des entreprises des évolutions en ce sens. Ce matin, la commission des finances interrogeait le

Afin de conserver la souplesse de son application, le projet de loi n'introduit pas de définition rigide de l'intérêt social, mais tend plutôt à en consacrer la notion dans la loi. Les sociétés ne sont pas gérées en vue de satisfaire

en prenant en considération ... » Quelle est la portée juridique de la « prise en considération » ? Je peux, quant à moi, considérer que, par moments, vous prenez en considération les amendements du Sénat. Cela peut arriver ! Mais il m'arrive assez souvent de penser que le Gouvernement ne les prend pas assez en considération. Vous allez pourtant, vous, avoir le sentiment que vous les prenez en considération.

Ensuite, comme pour toute obligation de moyens, il convient de se ménager la preuve que celle-ci a bien été remplie. Il s'agit de se prémunir contre toute décision judiciaire susceptible de juger que cette obligation n'a pas été mise en oeuvre. Tout ça est irréaliste pour une TPE ou une PME

Il est certain que ce pays manque de lois. Lorsque nous rencontrons des chefs d'entreprise, tous nous disent que le code du travail est vraiment trop mince, trop facile à appliquer ...

a voulu préciser les choses en tenant compte, justement, de l'évaluation des risques qui avaient été identifiés. Pour qu'il n'y ait pas de difficultés, la commission spéciale a clairement précisé que

est à Mme la secrétaire d'État. Il me semble qu'on ne peut pas ignorer- et je pense que vous ne l'ignorez pas, évidemment -que l'activité économique a un impact social et environnemental.

que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité », c'est simplement tirer le fil